J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion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

un outil de démocratisation de la culture, d'ouverture sur le monde, un lieu où nous venons partager des émotions, des rêves et où s'anticipent les mouvements de notre société. Hasard du calendrier, notre débat s'ouvre au moment où vient de s'achever le Festival de Cannes, qui contribue à faire rayonner le cinéma français à l'international. À cette occasion, comme chaque année, tous les acteurs du secteur se sont exprimés abondamment. Certains ont fait part de difficultés et d'inquiétudes qui seront certainement évoquées au cours de notre débat. Monsieur le ministre, vous-même vous y êtes largement exprimé et avez dessiné les contours d'un avenir possible. En France, le cinéma est un secteur stratégique qui, selon les chiffres du ministère, emploie plus de 100 000 personnes et représente 0,5 % de notre produit intérieur brut. brut. Rappelons que, selon les dernières statistiques du Centre national du cinéma, la France est le premier marché européen du cinéma en 2018, avec le niveau de fréquentation le plus élevé plus de 200 millions d'entrées pour la cinquième année consécutive. Cela démontre qu'il s'agit de la sortie culturelle préférée des Français. Le haut niveau de fréquentation des salles est lié à l'attractivité et à la diversité de l'offre de films, ainsi l'amélioration tant qualitative que quantitative des conditions de projection dans les salles. En cela, le développement des multiplexes depuis 1993 a certainement contribué à l'accroissement du nombre de spectateurs. Aujourd'hui, la France dispose du parc de salles le plus important et le plus dense d'Europe- le troisième du monde -, avec près de 6 000 écrans et un réseau encore bien ramifié dans les territoires. réseau d'exploitation, les films français rencontrent un important succès, avec une part de marché de près de 40 % et plus de 77 millions d'entrées, un chiffre en hausse de 1 % par rapport à 2017. Le secteur affiche une production importante de 300 films par an, y compris ceux qui sont coproduits

soit en termes de nombre d'entrées, de films produits ou de parts de marché. C'est, de toute évidence, le dispositif légal et financier mis en place par la puissance publique voilà fort longtemps qui a permis de soutenir le cinéma français et de préserver son dynamisme, sa créativité et sa diversité, y compris dans les périodes où la production nationale ne rencontrait pas le succès attendu. Le système français repose sur un principe vertueux consistant à faire remonter une partie des recettes de la diffusion vers la création, ce qui permet d'ailleurs de faire financer la création française

Il bénéficie également de crédits d'impôt, qui se sont révélés extrêmement efficaces, notamment le crédit d'impôt international, qui concerne les oeuvres dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. C'est un excellent soutien pour la filière cinématographique française.

de son environnement technologique, économique et financier, qui soulève des interrogations chez tous les acteurs. Ce bouleversement concerne la diffusion des contenus et les comportements des publics, qui évoluent également. Sous l'effet de la généralisation des technologies numériques, la circulation des oeuvres s'intensifie et les marchés s'ouvrent. On assiste donc à l'accélération des mouvements de concentration capitalistique des acteurs du secteur, qu'ils soient producteurs, distributeurs, exploitants ou diffuseurs. On peut dès lors craindre pour la survie de tout un tissu d'entreprises indépendantes qui deviennent peu rentables ou sous-capitalisées, mais qui restent essentielles pour la vitalité du cinéma français. Derrière le nombre rassurant de films produits, l'écart se creuse entre les grandes productions qui disposent de moyens importants et des films plus modestes qui restent peu de temps à l'affiche. Nous avons besoin des deux d'une diversité artistique représentant notre exception culturelle et d'un cinéma plus conquérant, qui assurera notre visibilité à l'étranger. L'arrivée de nouveaux acteurs dans le paysage audiovisuel et cinématographique- je pense aux grandes plateformes comme Netflix, Amazon et bientôt Disney,

durant cette période de 30,4 millions d'abonnés à plus de 139 millions. Elle est maintenant la plateforme la plus prolifique du monde. Le taux d'abonnement à Netflix au sein de la population française a plus que doublé

Concentration horizontale et verticale des acteurs mondiaux ; équilibre entre émergence en France d'acteurs puissants et exigence de diversité dans la création ; adoption par les géants du net de notre conception du financement de la création et du respect du droit d'auteur ; remise en cause de nos règles, désormais inadaptées à un marché ouvert et mondial

L'avenir du cinéma français, c'est le cinéma de Mati Diop, tantôt social et réaliste, tantôt onirique et mystique, un cinéma qui mélange les genres et surprend constamment c'est le cinéma ardent, percutant, furieusement authentique de Ladj Ly, dont l'empathie nous emmène au-delà des apparences, des clichés, des idées reçues sur nos quartiers ; c'est le cinéma résolument féministe de Céline Sciamma, qui chemine au plus près de l'émotion pour scruter l'étincelle qui déclenche la passion. Mati Diop, Ladj Ly, Céline Sciamma : tous les trois ont été récompensés samedi soir au Festival de Cannes. Cela me porte à croire que l'avenir du cinéma français est déjà là. Il est fait de leurs visages et de leurs noms. Il est fait de leur talent, de leur jeunesse, de leur audace folle, de leurs films merveilleux. Il est fait de ces voix qu'ils portent jusqu'à nous, et des regards qu'ils posent sur le monde : des regards singuliers, qu'ils nous font partager et qui changent un peu les nôtres. En tant que ministère des artistes, le ministère de la culture a une responsabilité : la responsabilité d'aider les cinéastes de demain à émerger, de leur permettre de s'exprimer, de créer, de se révéler, de rayonner. Le cinéma français nous a rappelé à quel point il est capable de rayonner. Il a rayonné à Cannes ; je viens de l'évoquer. En plus des trois films français présents au palmarès, deux autres sont des coproductions françaises. C'est sans précédent dans l'histoire du Festival Le cinéma français a rayonné aussi dans nos salles. En 2018, les films français y ont représenté plus de 40 % des entrées. À titre de comparaison, la part de marché du cinéma national est de 24 % en Allemagne, de 18 % en Espagne ou de 12 % au Royaume-Uni. C'est un succès d'autant plus significatif que la fréquentation de nos salles de cinéma s'est maintenue à plus de 200 millions d'entrées, pour la dixième année consécutive, soit quasiment le double du nombre annuel d'entrées en Allemagne. Ces chiffres sont éloquents : la France est une nation de cinéphiles. Ainsi, 65 % de nos concitoyens se rendent au cinéma au moins une fois par an, ce qui en fait la sortie culturelle la plus populaire. Et ils s'y rendent partout sur le territoire : une salle sur deux se trouve dans une commune de moins de 10 000 habitants

Grâce à la réforme des trois crédits d'impôt dédiés à la production cinématographique et audiovisuelle, la France est redevenue attractive pour les tournages. Le taux de délocalisation des dépenses des films français a été divisé par deux. Plus de 500 millions d'euros de dépenses de tournage supplémentaires ont été effectuées dans notre pays chaque année. Enfin, 15 000 emplois ont été créés. Aujourd'hui, la filière du cinéma et de l'audiovisuel représente 0,8 % du PIB et 340 000 emplois. Ces chiffres, ces succès, ce rayonnement du cinéma français ne viennent pas de nulle part. Ils sont le fruit d'une politique publique volontariste engagée par la France voilà soixante-dix ans et patiemment poursuivie depuis, une politique en faveur du cinéma qui a doté la France d'un modèle unique au monde, appréhendant et incluant tous les maillons de la filière : auteurs, producteurs, distributeurs, ainsi que l'ensemble des diffuseurs, qu'il s'agisse des salles de cinéma, des éditeurs de vidéos, des chaînes de télévision, des fournisseurs d'accès à internet, plateformes de téléchargement à l'acte ou par abonnement. Pour permettre au cinéma français de briller demain davantage encore, il faut défendre ce modèle. Pour cela, il faut l'adapter aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain. J'en vois trois. Le premier enjeu est celui de l'égalité et de la diversité. Dans le cinéma, comme dans trop d'autres domaines, nous sommes encore loin de l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes toutefois sur la bonne voie. Cette année, treize réalisatrices ont été sélectionnées au Festival de Cannes, toutes sélections confondues. C'est un record.

Un quart des films soutenus depuis le début de cette année ont pu en bénéficier. Il faut aller encore plus loin sur la question de l'égalité, comme sur celle de la représentation de la diversité. Trop souvent, les écrans ne montrent qu'une partie de notre société ; trop souvent, ils occultent sa diversité. Or, pour que le cinéma parle à tous, il faut qu'il parle de tous. C'est pourquoi le CNC organisera de nouvelles assises à la rentrée prochaine, sur le thème de la diversité. J'en suis convaincu, pour continuer à attirer le public dans les salles, le cinéma doit s'emparer encore davantage de ces questions. Le deuxième enjeu est celui de la régulation des géants du numérique. Ce n'est pas parce que ce sont des géants qu'ils peuvent échapper à toute régulation. Ils nous disent en être conscients,

Mais ils doivent également coopérer sur d'autres sujets et contribuer, comme les autres acteurs, au financement de la création, à la diversité culturelle et au respect des droits des auteurs. Il nous faut donc intégrer les acteurs du numérique à notre modèle de financement de la création audiovisuelle et cinématographique. Cela passe d'abord par un rééquilibrage du poids de la fiscalité et de la réglementation entre les entre les diffuseurs « historiques » du cinéma et les nouveaux entrants que sont les plateformes numériques. C'est un enjeu d'équité, de neutralité technologique et économique et de simplification. En matière fiscale, un premier pas a été franchi avec la mise en place, en 2018, d'un prélèvement de 2 % sur le chiffre d'affaires des plateformes de diffusion, qu'elles soient gratuites ou payantes. Mais nous souhaitons aller plus loin, ce qui contribuera à consolider les ressources du CNC dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020. L'intégration des nouveaux acteurs à notre modèle passera aussi par le projet de loi qui transposera la directive « services des médias audiovisuels », ou SMA. Il s'agira d'une loi ambitieuse. Elle sera ambitieuse en matière d'obligations de diffusion : la directive SMA prévoit que les plateformes proposent au moins 30 % d'oeuvres européennes. Non seulement c'est un minimum, mais nous ferons en sorte que les oeuvres européennes soient mises en valeur dans les recommandations personnalisées. La loi sera ambitieuse aussi en matière d'obligations d'investissement. Enfin, elle le sera pour garantir l'indépendance de nos entreprises de production par rapport aux plateformes. L'arrivée de ces nouveaux financeurs, riche en potentialités, ne doit pas transformer notre filière en une simple activité de sous-traitance. La transposition de la directive doit également permettre d'inscrire dans la loi les règles de transparence sur les données d'exploitation des oeuvres qui s'appliqueront à tous les diffuseurs, plateformes comprises. C'est indispensable pour s'assurer du respect du droit d'auteur et des droits voisins. Plus généralement, cette transparence est la base de la relation de confiance entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. La loi offrira enfin l'occasion de renforcer la lutte contre les sites pirates, notamment de piratage « en flux » et de téléchargement direct. Le dernier enjeu de l'adaptation de notre politique est le nécessaire renforcement des entreprises de production et de distribution, parce que pérenniser l'exception culturelle, ce n'est pas seulement aider à la création des oeuvres. C'est aussi permettre à la production et à la distribution d'attirer de nouvelles sources de financement privé et de mieux se structurer ; je pense en particulier à la production indépendante. Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux que l'avenir du cinéma français soit radieux. Pour cela, notre cinéma devra être plus paritaire, plus représentatif de la diversité. Il devra intégrer les acteurs du numérique à son modèle de financement, et sa production et sa distribution devront être renforcées. Voilà quelques-uns des combats que nous aurons à livrer. Pour les mener, vous pouvez compter sur ma détermination. La France est la patrie du cinéma, et elle le sera encore demain ! Nous allons maintenant chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

rien ne sera possible sans un partenariat étroit entre l'État et les territoires, rien ne sera efficace sans un travail en confiance avec les acteurs et les élus locaux, qui accompagnent au quotidien les dynamiques d'innovation et de développement économique. C'est une des leçons qu'il faut tirer du grand débat national. Je me félicite que le Président de la République ait appelé à un nouvel « acte de décentralisation ». Ce nouvel acte de décentralisation, il faut maintenant le traduire le plus rapidement possible dans les faits, car des dynamiques locales particulièrement remarquables sont à l'oeuvre et doivent être encouragées et soutenues. C'est le cas

un lieu exceptionnel, avec 300 hectares de terrains qui ont d'ores et déjà accueilli des décors extérieurs destinés au tournage de films, notamment, nominé pour le César 2019 du meilleur décor. Aujourd'hui, le succès du Backlot 217 est le fruit d'un partenariat actif entre Coeur d'Essonne agglomération et la société TSF Studios, acteur cinématographique majeur en France et en Europe depuis 1979. Cette dernière souhaite désormais investir 14 millions d'euros pour construire 14 000 mètres carrés de plateaux, et 10 hectares de terrains supplémentaires pourraient être proposés afin de réaliser ce projet.

La fréquentation des salles a même baissé de 4,3 %. Dès lors, ceux-là mêmes qui étaient les apôtres de l'ouverture, du multiculturalisme et de la diversité dans tous les secteurs de l'économie sont pris de panique devant le scénario possible de la perte, pour certains, de juteux bénéfices, et, pour d'autres, de leur emploi. On n'hésite pas à brandir l'« exception culturelle française », sorte de préférence nationale à peine déguisée ... Au-delà de l'ironie et de l'hypocrisie, convenons que le cinéma français est une exception. Avant d'être une industrie, il est un art. Si, outre-Atlantique, le cinéma rapporte, en France, il apporte il apporte des émotions aux spectateurs grâce à des scénaristes de génie, des metteurs en scène exceptionnels, des acteurs qui, pour certains, sont devenus des monstres sacrés, au point que le calamiteux Festival de Cannes a été obligé cette année de rendre un hommage au très politiquement incorrect Alain Delon

Attaqués par le libéralisme consumériste et par le prêt-à-penser, qui se traduit par le prêt-à-filmer, le prêt-à-jouer, les Français se détournent d'un cinéma subventionné, politisé, aseptisé, qui ne les fait plus rêver, qui ne les divertit plus, dans lequel ils ne se reconnaissent plus.

Particularité française, les salles d'art et d'essai maintiennent un lien social et une diversité culturelle très précieux. On a besoin, plus que jamais, de films qui offrent un point de vue singulier, complexe et sensible sur le monde contemporain ou présentent de nouveaux imaginaires. Ces films sont cependant de plus en plus difficiles à produire. et essai » regroupe 1 182 établissements, soit près de la moitié des cinémas hexagonaux. Aux antipodes de la plupart des grands réseaux, qui se financent en visant un large public avec des, ces petits exploitants font parfois vivre les derniers lieux culturels de proximité implantés dans des zones rurales. Ils sont donc de vrais vecteurs

Nombre d'entre eux sont aidés par les municipalités ou les intercommunalités. Un cinéma sur deux est lié à une collectivité. Ils subissent donc les effets cumulés de la baisse des dotations budgétaires et de la réforme territoriale.

de part de marché pour les longs-métrages, l'horizon du cinéma français semble plutôt au beau fixe. Mais, comme le titrait la semaine dernière, n'est-il pas un malade bien portant ? En effet, son financement se dégrade peu à peu, d'où une fragilisation d'un secteur qui représente pourtant à la fois un art et une industrie essentiels pour notre pays, reconnus et appréciés dans le monde entier. Il devient donc urgent de réinventer l'architecture du financement du cinéma français pour en préserver le dynamisme, la qualité et la richesse. Certains prônent le développement du financement privé : pourquoi pas, mais cela ne doit pas conduire à faire de la rentabilité le critère principal de sélection, au détriment de la diversité de notre septième La politique publique d'aide au cinéma mérite d'être modernisée pour assurer une meilleure diffusion des films auprès du public et un meilleur soutien aux talents. Ne convient-il pas dès lors d'avoir avant tout une approche globale, en mettant autour de la table tous les acteurs concernés pour réfléchir à l'avenir du cinéma français ? L'Union européenne a toute sa place dans ce tour de table. D'une part, parce qu'elle finance depuis 1991 de nombreux projets audiovisuels, notamment au travers du programme Media, dont le budget n'a cessé d'augmenter, même s'il reste insuffisant, jusqu'à atteindre 1 milliard d'euros pour la D'autre part, parce que la bataille est à mener sur de nombreux fronts ; je pense notamment à la révolution numérique et aux grandes plateformes de diffusion étrangères, qui doivent davantage participer au financement du cinéma français et européen. Dès lors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour renforcer la défense et le financement du cinéma français au niveau européen, notamment en allant plus loin que la directive « services de médias audiovisuels » La France, terre de cinéma, va-t-elle prendre le sur tous ces sujets ? Comment comptez-vous rallier l'ensemble de l'Europe à notre conception de l'exception culturelle, pour préserver le cinéma français ? La parole

pour les industries culturelles et créatives. Doté de 225 millions d'euros, il s'ajoutera aux dispositifs d'aide et de crédit d'impôt pour structurer financièrement les entreprises, notamment de la production, qui ont besoin de capitaux pour se développer et investir dans le préfinancement des oeuvres ou l'acquisition d'oeuvres.

Depuis sa création, elle a émis plus de 10 millions d'avertissements, pour des résultats appréciables : sur dix personnes averties, six prennent des mesures pour éviter tout renouvellement d'actes de piratage. Cependant, il devient nécessaire d'adapter le cadre existant, en raison de l'évolution des pratiques. En effet, la Hadopi surveille les internautes qui téléchargent « de pair à pair », mais cette technique est de moins en moins utilisée. Près de 80 % du piratage en France se fait maintenant le, qui représente 66 % des actes illégaux, ou par téléchargement direct, à l'abri des radars de la Hadopi, l'accès à l'adresse IP de l'abonné étant impossible. Par ailleurs, l'écosystème illicite se complexifie, avec l'apparition d'une pluralité d'acteurs intervenant en amont ou en aval des pratiques de piratage pour mieux les organiser, ainsi que le perfectionnement des mesures de contournement. Pour faire face à ces nouvelles pratiques, votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait indiqué des pistes de réforme : extension des prérogatives de la Hadopi, établissement d'une liste noire des sites illicites, blocage ou déréférencement des sites, responsabilisation des plateformes numériques Vous souhaitez, monsieur le ministre, traiter le sujet du piratage au travers d'un grand projet de loi sur l'audiovisuel, mais la présentation de celui-ci est régulièrement reportée et vous l'avez à peine évoqué dans votre propos liminaire. Pourriez-vous nous préciser quelles dispositions vous comptez proposer, et selon quel calendrier ? Bravo ! La parole

d'accès à internet et les moteurs de recherche doivent bloquer et déréférencer les sites pirates à leurs frais, quand l'ordre leur en est donné par un juge.

Jean Gabin, sans doute le plus parisien des acteurs français, avait une conception très tranchée de ce qui pouvait faire un bon film : premièrement, une bonne histoire ; deuxièmement, une bonne histoire ; troisièmement, une bonne histoire. Sans le rejoindre totalement, tant j'aime les films dits « de mise en scène », je voudrais tout de même que ce débat soit l'occasion de rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui rendent possibles ces émotions, quelle que soit la forme sous laquelle on regarde les films, bref à celles et ceux qui écrivent le cinéma, car le cinéma s'écrit aussi.

Comme l'économie dans son ensemble, le monde du cinéma est traversé par des évolutions qui peuvent parfois préoccuper les scénaristes français, à commencer par la montée en puissance d'opérateurs nouveaux- Netflix ou Amazon, pour ne pas les nommer -, qui créent leurs propres viviers de scénaristes. Il faut également garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses façons d'exercer ce métier de scénariste, par exemple en se lançant dans une création ou en adaptant une oeuvre littéraire.

se fait souvent à plusieurs mains : moins de 5 % du budget d'une oeuvre est consacré aux dépenses d'écriture et la rémunération complémentaire sur l'amortissement du film est encore faible pour les scénaristes de cinéma.

et évaluer les besoins du secteur en matière de services aux scénaristes et de formation à l'écriture. Plus largement, j'ai pris la décision de créer une mission, présidée par Bruno Racine, associant des universitaires, des sociologues et, évidemment, des professionnels du secteur, afin de réfléchir à la place des artistes-auteurs dans la société. Cette mission prospective doit nous permettre

qui ont peut-être contribué à une augmentation de la fréquentation cinématographique, mais qui contribuent aussi à la dévitalisation des centres-villes. Chacun sait à quel point nombre de nos nombre de nos territoires se sentent aujourd'hui abandonnés. La raréfaction de l'offre culturelle y est, je le crois, pour quelque chose, d'autant que le cinéma a toujours occupé une place particulière dans l'accès à la culture. Plusieurs d'entre nous ont rappelé à juste titre que c'est la sortie culturelle la plus populaire.

Ce sont pourtant ces salles qui font du cinéma une pratique culturelle à part entière, qui sont souvent les premières à oeuvrer pour une diversité de films projetés et à mettre en place des activités culturelles et éducatives autour du cinéma.

des auteurs reconnus et récompensés dans les grands festivals, grâce à la signature d'engagements de diffusion par les distributeurs. Nous travaillons à un futur plan d'action 2019-2021 pour les salles d'art et d'essai. La

Le Gouvernement a fait un choix très clair : celui de rééquilibrer les contraintes entre les acteurs historiques et les nouveaux entrants, d'augmenter, pour les

l'Europe ont lancé l'appel suivant pour inciter nos concitoyens à voter lors des élections européennes : « L'Europe, nous nous efforçons de la décrire avec la délicatesse des images et un langage plus accessible à tous les peuples qui la composent. [ ...] Une Europe libre et démocratique, c'est aussi une Europe de la libre pensée et et de la liberté d'expression. » Au-delà du vote, la préoccupation de ces grandes figures est bien celle de l'Europe de la culture, qui peine à exister, à se fédérer. Dans ce contexte, je souhaite vous faire une proposition, que j'ai déjà eu l'occasion de formuler

la mise en place d'un fonds de 225 millions d'euros, opéré par Bpifrance et destiné à aider les entreprises du secteur de la création. Pourquoi ne pas consacrer une partie significative de ce fonds à l'amorçage d'une grande plateforme européenne, respectueuse de nos règles en matière de production et de diversité ? Cela permettrait peut-être de lutter enfin à armes égales avec les plateformes extraeuropéennes. Un tel outil aurait les moyens de produire des films, des séries et des documentaires, la créativité en la matière étant la meilleure garantie du succès.

capitaux. La présence des contenus français et européens sur les plateformes est un enjeu

privés et publics dans la structuration d'une offre numérique de mise à disposition des contenus français et européens. Il y a là un véritable enjeu de souveraineté et de défense

Morin-Desailly, pour la réplique. Certains pensent que nous avons déjà perdu la bataille des tuyaux et des outils, et que nous sommes maintenant dans la bataille des contenus. Je ne suis pas complètement d'accord avec cette vision minimaliste ; au contraire, soyons volontaires. Ce que l'on attend de l'État actionnaire, c'est qu'il fédère les acteurs et qu'il donne le ton,

est à Mme Laure Darcos. Monsieur le ministre, j'ai cru comprendre que Netflix venait de s'offrir les droits de deux films primés au Festival de Cannes. En acquérant les droits de ces longs-métrages, cette plateforme de vidéo à la demande contourne les règles du Festival, qui a pour principe de refuser les projets n'ayant pas vocation à être diffusés en salle. Ce contexte témoigne de la montée en puissance des plateformes de vidéo à la demande : Netflix, Amazon Prime, Disney Fox et, bientôt, Apple. La directive européenne « services de médias audiovisuels », adoptée en 2018, a établi la possibilité d'imposer à ces plateformes étrangères des obligations d'investissement dans des oeuvres européennes et françaises, sur le fondement de leur chiffre d'affaires réalisé en France. Au regard du décret du 12 novembre 2010 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande, qu'il conviendrait de réécrire, Netflix, Amazon Prime et Disney Fox devraient consacrer entre 12 % et 15 % de leur chiffre d'affaires annuel réalisé en France à la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises. Pour Netflix, cela représenterait un investissement annuel compris entre 55 millions et 90 millions d'euros dans des oeuvres européennes, et entre 40 millions et 75 millions d'euros dans des oeuvres françaises. Ces chiffres sont élevés et pleins de promesses pour le secteur. Compte tenu de la différence de plus en plus ténue entre les chaînes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande avec abonnement, il serait judicieux, de mon point de vue, de mettre en place deux réformes. La première consisterait à unifier les taux d'investissement dans les oeuvres à partir d'un certain chiffre d'affaires, sans distinction entre services linéaires et non linéaires la seconde consisterait à imposer qu'une part significative de cet investissement se fasse en préachat, c'est-à-dire au moment de la constitution du budget de l'oeuvre. Ces propositions peuvent-elles retenir votre attention, monsieur le ministre ? Par ailleurs, entendez-vous mettre fin à la différence existant entre les investissements réalisés dans le cinéma et ceux qui

obligations, les mêmes règles d'investissement et d'exposition, que les acteurs historiques ; en même temps, nous devons les accueillir comme il se doit : ce sont des acteurs qui viennent investir en France dans des contenus, il ne faut pas

jouissent de l'estime et de la reconnaissance de l'ensemble de la société pour leur création, beaucoup se retrouvent dans une situation sociale particulièrement délicate, pour ne pas dire précaire. eux ont un revenu équivalent au SMIC, et un artiste-auteur sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. En d'autres termes, si l'acte de création est valorisé dans la société, la rémunération qui y est attachée est parfois dérisoire.

la retraite. Le code de la sécurité sociale dispose que, pour les auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, les producteurs prennent en charge une fraction de la cotisation versée à la caisse de retraite complémentaire, fraction dont le niveau est défini par décret. Or le texte réglementaire est attendu depuis environ deux ans. Ainsi, en l'état, la loi n'est pas pleinement appliquée, et une charge financière pèse sur les auteurs de l'audiovisuel et du cinéma.

de Bong Joon-ho. Le Festival avait alors été surpris que Netflix ne se plie pas à sa règle voulant que tout film sélectionné en compétition officielle sorte en salles en France. Néanmoins, cette règle est sûrement obsolète

en salles, ce qui lui a permis de concourir à Cannes. Il a même remporté la Palme d'or, ce qui prouve que le mode de diffusion ne détermine pas la valeur d'une oeuvre ; un film vaut par sa forme. Du reste, cette exigence de sortie reste, cette exigence de sortie en salles ne vaut pas pour d'autres rendez-vous internationaux du cinéma, tels que le festival de Berlin ou la Mostra de Venise, qui a d'ailleurs couronné, en 2018, un film distribué par Netflix,. Netflix,. Les dirigeants du Festival de Cannes arguent que Netflix n'est pas accessible à l'ensemble des Français, contrairement aux salles de cinéma, mais l'abonnement à Netflix coûte 11 euros par mois, pour un écran que l'on peut regarder à plusieurs, quand on le souhaite et autant de fois qu'on le

fait que l'on s'achemine vers un décalage croissant entre le cinéma subventionné et la réalité de la consommation des films. Netflix est une menace pour le cinéma français, il a dépassé la barre des cinq millions d'abonnés en France, mais, au fond, le cinéma français et la plateforme de sont peut-être complémentaires. Le cinéma français peut-il survivre à

davantage au financement et à l'exposition des films. Il sera alors temps de réfléchir à une éventuelle évolution supplémentaire de la chronologie des médias.

de la politique budgétaire du Gouvernement.

bien. Alors même que la France, patrie des frères Lumières et de Georges Méliès, est le berceau du cinéma, cet art majeur et populaire, qui opère la synthèse de tous les arts audiovisuels, ne dispose pas dans notre pays d'un musée d'envergure internationale. Afin de remédier à cette carence, la mairie de Cannes vient de lancer la création d'un musée international du cinéma et du festival. Une telle démarche est parfaitement légitime pour la ville qui accueille depuis soixante-dix ans le plus grand festival de cinéma et le premier événement culturel du monde. En outre, Cannes et sa communauté d'agglomération, Cannes Pays de Lérins, ont engagé un ambitieux programme pour devenir le territoire d'excellence de l'économie créative, avec le développement d'une filière complète de l'audiovisuel, incluant la formation de créateurs, la mise en place d'un campus universitaire dédié aux métiers de l'écriture, l'accompagnement d'entreprises du secteur audiovisuel, la création de contenus, la distribution et la diffusion d'oeuvres culturelles et l'organisation d'événements afin d'en assurer la promotion.

Parallèlement, grâce à une politique volontariste, le nombre de prises de vues et de tournages sur le bassin cannois est passé de 128 en 2015 à 562 en 2018. 2018. En parfaite cohérence avec cette stratégie territoriale axée sur le développement de l'économie créative et audiovisuelle, Cannes se propose d'accueillir toute l'année le cinéma du monde d'hier, d'aujourd'hui et de demain, en hébergeant sur son territoire un musée international du cinéma et du Festival de Cannes. Soutenir l'institution d'un tel équipement culturel majeur en province montrerait la volonté forte du Gouvernement de conduire une politique affirmée de décentralisation culturelle, comme cela s'est fait avec le Louvre-Lens ou le Centre Pompidou-Metz. Monsieur le ministre de la culture, quels efforts d'accompagnement l'État est-il prêt à consentir pour permettre à ce projet, lancé par le maire de Cannes, de disposer des ressources, publiques et privées, émanant de l'industrie du cinéma, nécessaires à sa réalisation ?

bougeaient ! Claude Chabrol défendait toutes les formes de cinéma. Or on constate aujourd'hui un écart de plus en plus important entre les films abondamment financés et les petites productions qui ont du mal à boucler leur budget. La puissance publique a encore la faculté de garantir l'exception culturelle française. À ce titre, il serait utile d'améliorer l'intervention du CNC en appui au développement économique de l'industrie du cinéma,

une politique publique a toujours vocation à être analysée, évaluée et, le cas échéant, réorientée. Ce que vous dites est tout à fait juste : nous devons veiller à ce que les politiques d'accompagnement de la production et de la création cinématographiques n'oublient pas

Je voudrais terminer sur une note optimiste, car je crois qu'il y a lieu de l'être. La capacité de résistance du cinéma résulte en partie de sa nature même, caractérisée, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre, par une émotion partagée collectivement en salle. Robert Desnos disait : « Ce que nous demandons au cinéma, c'est ce que l'amour et la vie nous refusent, c'est le mystère, c'est le miracle. » Cette demande existe sans doute toujours aujourd'hui, et pour longtemps encore.

La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, questions d'actualité au Gouvernement. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

socialiste et républicain. Ma question, à laquelle je souhaite associer mon collègue Martial Bourquin, s'adresse au Premier ministre. La Bourgogne-Franche-Comté est la première région industrielle du pays au regard de la part des salariés de l'industrie dans la population active. C'est une fierté pour tous ses habitants et c'est un atout pour notre pays. Ce matin, la direction de General Electric a reçu les représentants syndicaux pour leur annoncer un plan de restructuration. Il prévoit la suppression de plus d'un millier d'emplois dans le Territoire de Belfort, sur les sites GE de Belfort et de Bourogne. C'est un quart des effectifs de GE que la direction souhaite rayer d'un trait de plume. C'est un coup de massue pour toute la population. Pourtant, à la suite du rachat de la branche énergie d'Alstom, le même groupe GE nous promettait la création de 1 000 emplois. Beaucoup attendaient mieux de M. Macron, qui a surtout su négocier le calendrier de ce plan social, annoncé au lendemain des élections européennes. Eh oui ! M. Montebourg avait mis en place des garanties lors de la vente d'Alstom. Elles alimenteront un fonds précieux de réindustrialisation, à hauteur de 50 millions d'euros. Toutefois, ce fonds n'est toujours pas opérationnel, malgré l'insistance des collectivités locales. Aujourd'hui, l'annonce de GE constitue une nouvelle rupture, qui appelle une réponse forte de la part de l'État. GE doit préserver davantage d'emplois et de savoir-faire, diversifier son activité sur les sites de Belfort et de Bourogne, mais aussi remettre la main à la poche Monsieur le ministre, quels sont vos objectifs en termes de réduction du nombre d'emplois supprimés ? Êtes-vous prêt à exiger le doublement de l'amende due par GE ? Comment allez-vous associer les élus locaux du territoire, qui forment une union sacrée, pour assurer un avenir à l'industrie régionale ?

C'est un coup dur pour les salariés de GE. Il résulte tout simplement de l'effondrement des commandes de turbines à gaz. Vous connaissez parfaitement le dossier : 100 turbines à gaz avaient été commandées à GE Belfort en 2008, contre 29 aujourd'hui, et les perspectives pour les années à venir ne sont pas bonnes. seront-elles plus ouvertes à compter de 2040, lorsque les usines à charbon auront fermé, mais, dans l'intervalle, il faut trouver d'autres activités. Mon objectif principal est de trouver de nouveaux débouchés industriels pour les salariés de GE à Belfort.

nécessaires sont présentes -, mais aussi dans le démantèlement des centrales nucléaires et dans les grands carénages. Dans tous ces domaines, qu'il s'agisse de l'aéronautique, du nucléaire ou de l'hydrogène, les salariés ont les compétences et les qualifications nécessaires pour réinventer un avenir industriel sur le site de Belfort.

Nous devons en tirer les enseignements, afin d'apporter immédiatement des réponses claires et concrètes à leurs attentes légitimes. Force est de constater que la fracture territoriale qui se creuse depuis déjà de nombreuses années est désormais indiscutable. Le résultat de ces élections européennes marque une nouvelle accentuation de la différence entre le vote urbain et le vote rural. Nous n'en sommes pas surpris, car les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La disparition des services publics et le désengagement de l'État sont bien réels. J'ai pu observer que, partout où le lien social est développé et vivant, la progression des populistes a été freinée. Dimanche soir, le Gouvernement a indiqué que l'acte 2 du quinquennat allait commencer. Monsieur le Premier ministre, quelle lecture faites-vous des résultats et quelles mesures comptez-vous prendre pour résorber la fracture territoriale ? En tant que sénateur de la Meuse, je sais que vous pourrez vous appuyer sur les élus locaux pour relever les défis territoriaux.

C'est la raison pour laquelle, sous l'autorité du Premier ministre, un certain nombre de chantiers ont d'ores et déjà été lancés, en particulier une mobilisation nationale pour l'emploi dans les territoires, qui permettra aux partenaires sociaux et aux collectivités locales de s'unir

Nous en arrivons aujourd'hui à une véritable pénurie dans les officines, ce qui contraint les patients à se livrer à une surréaliste chasse au trésor. Pouvez-vous nous expliquer précisément comment cette situation incroyable et inacceptable a pu

En effet, dès que l'ANSM a été informée, début mai, de l'existence de tensions en matière d'approvisionnement en corticoïdes, elle a immédiatement convoqué les fabricants afin qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'accès des patients à ces médicaments dans les plus brefs délais. Cela s'est traduit par la mobilisation par les fabricants de stocks permettant de garantir la couverture des besoins des patients. L'ANSM a également régulièrement échangé avec les représentants d'associations de patients et les professionnels de santé pour partager les informations à sa disposition.

ou injectables. Le retour à une disponibilité normale de ces médicaments dans les pharmacies d'officine ou hospitalières est attendu d'ici à la fin du mois de juin. Entre-temps, l'ANSM maintient son dispositif de suivi renforcé. Un tableau de la disponibilité des différentes spécialités par dosage est public et consultable sur le site de l'agence. Nous faisons le choix d'une gestion transparente de ces dossiers. Si les autorités n'ont pas tardé à réagir, il n'en demeure pas moins que la situation actuelle, en termes de rupture de médicaments, n'est pas acceptable pour les Français. Mme la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, présentera dans quelques jours un plan d'action destiné à éviter la pénurie de médicaments et à avoir une visibilité sur la gestion des stocks. La parole

Ainsi, un collectif de 500 chercheurs a dénoncé l'omerta qui règne sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu universitaire. J'apprends que ces affaires sont censées être traitées selon des procédures disciplinaires laissées à la discrétion du président de l'établissement ou de la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont la compétence et la probité ont été ouvertement mises en cause par deux articles de datés du 20 mai dernier. dernier. Le nombre de procédures et les sanctions appliquées sont dérisoires au regard de l'ampleur du phénomène. Les victimes sont entendues comme simples témoins ou ne sont carrément pas auditionnées, et elles ne disposent d'aucun mécanisme d'appel, contrairement aux agresseurs La procédure disciplinaire est une première étape importante pour la victime, qui peut ainsi être reconnue comme telle. Cela permet surtout d'arrêter immédiatement les agissements des agresseurs. Mais encore faut-il que procédure disciplinaire il y ait madame la ministre ! Vous le savez d'ailleurs, pour avoir annoncé l'ouverture de cellules de veille dans chaque université et proposé une large campagne de formation du personnel des Crous sur ces questions. Crous sur ces questions. Nous sommes fin mai 2019 : combien d'universités sont-elles dotées de cellules de veille ? Comment répondre aux attentes des victimes qui se heurtent à des procédures disciplinaires opaques et apparemment peu rigoureuses ?

Madame la ministre, les violences sexuelles, outre qu'elles détruisent durablement leurs victimes, ont un coût très lourd pour la société en termes de santé publique. Éradiquer ce fléau où qu'il se manifeste -famille, école, église, université

Le groupe Renault a annoncé, ce lundi 27 mai, avoir reçu une proposition de Fiat Chrysler Automobiles, FCA, concernant une potentielle fusion à parité. Renault a fait savoir que son conseil d'administration avait décidé d'examiner avec intérêt l'opportunité d'un tel rapprochement, qui, en cas de fusion, ferait de la nouvelle entité le troisième groupe automobile mondial, et même le premier en y ajoutant le tandem Nissan-Mitsubishi.

Les deux groupes sont bien placés sur des marchés complémentaires et espèrent aussi se renforcer sur de nouveaux secteurs géographiques. Le secteur automobile est confronté à des défis majeurs, le véhicule autonome et la voiture électrique exigeant des investissements massifs. Seuls de grands ensembles industriels seront en capacité d'effectuer les investissements qui assureront les emplois de demain dans l'industrie automobile. Cette fusion peut permettre à Renault-Nissan et à et à FCA de constituer un champion européen compétitif, avec des bases européennes. En matière de véhicules, c'est une nouvelle ère qui commence, avec la fin programmée des moteurs thermiques en France d'ici à 2040. À cet effet, Renault a déjà investi l'an dernier un milliard d'euros dans les usines de Douai et de Maubeuge, où est fabriquée la Kangoo électrique. Le groupe fusionné pourrait devenir le leader mondial dans un secteur en pleine évolution, avec un fort positionnement dans les nouvelles technologies. cette fusion peut permettre de relever les défis de demain dans le secteur automobile, elle soulève aussi des questions. J'en vois deux, essentielles : ce projet de fusion représente-t-il une menace pour l'emploi et les intérêts de l'État ? Sa mise en oeuvre aurait-elle une incidence sur l'alliance Renault-Nissan ?

sur cette question, au cours duquel nous avons réaffirmé notre volonté de renforcer l'alliance entre Renault et Nissan. Jean-Dominique Senard est aujourd'hui au Japon pour engager les discussions avec nos partenaires japonais.

Si les métiers d'aide-soignant et d'auxiliaire de vie souffrent d'une sévère désaffection depuis plusieurs années déjà, s'y ajoute désormais une véritable crise des vocations chez les infirmiers. Les services hospitaliers rencontrent en effet de grandes difficultés à recruter et, surtout, à garder leur personnel, et les écoles d'infirmières peinent à se remplir. Les causes sont multiples, mais la question d'une juste rémunération Nous pouvons voter toutes les lois de réorganisation possibles, en l'absence d'un financement à la hauteur des enjeux et d'une reconnaissance de nos personnels soignants, le système se tend et risque la rupture. J'en veux pour preuve le fait que de très nombreux établissements peinent à assurer un exercice optimal de leur activité et sont souvent contraints de recourir à des intérimaires, bien plus coûteux.

franchissent chaque jour la frontière pour aller travailler. Un article récent d'un grand quotidien en fait état et pointe des conditions générales d'exercice bien plus favorables chez nos voisins, en particulier au Luxembourg, le salaire moyen d'une infirmière en début de carrière est quasiment le double de ce qu'il est en France. La quasi-totalité de nos voisins proposent également des rémunérations plus élevées.

et concrètes de nature à les rassurer. Quelles dispositions entendez-vous prendre, y compris à une échelle transfrontalière, pour remédier au manque d'attractivité de ces métiers ?

le Gouvernement partage votre préoccupation quant à la moindre attractivité financière des postes ouverts en France. Les infirmiers, comme les aides-soignants et les auxiliaires de vie, jouent un rôle central dans notre système de santé et sont indispensables, au quotidien, au fonctionnement de nos établissements de santé. Aussi cette situation ne peut-elle que nous préoccuper.

Les établissements de santé de ces régions frontalières ont déjà pris des initiatives tendant à la création d'observatoires transfrontaliers des personnels de santé. Ces expériences conduites entre les différents pays

pour les infirmiers de la fonction publique hospitalière engagés dans un protocole de coordination. Parallèlement à cette réflexion, les travaux conduits par le ministère pour revaloriser les métiers se poursuivent. Le sixième avenant de la convention des infirmiers libéraux a été signé fin mars avec l'assurance maladie.

voilà une présentation rapide du projet de mine « Montagne d'or » en Guyane. Depuis 2014, le Président Macron est un fervent partisan de ce projet, mais les peuples autochtones, les ONG et 70 % du peuple guyanais dans son ensemble y sont opposés. À quinze jours du scrutin européen, et avant de recevoir le chef amérindien Raoni,

celle du ministre de la transition écologique et solidaire, selon lequel le projet ne se fera pas, comme l'a répété la porte-parole du Gouvernement, acculée par de nombreuses questions sur un plateau de télévision, dimanche soir ? Si nous disons « chiche » à une réforme du code minier instaurant l'interdiction de

Ce projet est incompatible avec les exigences de protection de l'environnement, de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique qui sont défendues par ce gouvernement et exigées par les Français. Je le

Il y a deux mois, le gouvernement auquel vous appartenez affirmait suivre avec la plus grande attention la réorganisation de GE. Il expliquait souhaiter accompagner le développement d'activités nouvelles, telles que l'aéronautique, le grand carénage ou encore l'hydrogène, auquel je crois beaucoup. Plus inquiétant, le Gouvernement excluait d'office son soutien aux projets liés aux énergies fossiles, notamment le gaz, comme l'exprimait votre secrétaire d'État dans cet hémicycle le 4 avril dernier. Vous avez même personnellement affirmé qu'il n'y avait pas d'avenir pour le marché des turbines à gaz. C'est aujourd'hui que la nouvelle tant redoutée est tombée. Une catastrophe industrielle pour mon département et pour le nord de la Franche-Comté : 1 044 emplois seront supprimés par General Electric à Bourogne, à Boulogne-Billancourt et à Belfort, site qui va perdre 985 de ses salariés ! Un salarié sur quatre sera touché. Des drames s'annoncent ; des familles vont se trouver en difficulté. Mes premières pensées vont, bien entendu, aux femmes et aux hommes touchés par ce tsunami industriel. Monsieur le ministre, l'heure n'est plus aux petits arrangements calendaires, comme avec cette annonce que GE a opportunément retardée jusqu'au lendemain des élections européennes. Les salariés ont besoin de réponses concrètes. Quels choix stratégiques le Gouvernement met-il en oeuvre pour le redressement de l'industrie belfortaine ? Quels efforts de réindustrialisation êtes-vous en mesure de porter pour ce territoire ? Excluez-vous, oui ou non, les projets liés aux énergies fossiles ?

les salariés, tous ceux qui travaillent sur le site de GE à Belfort et l'ensemble des élus locaux, que j'ai rencontrés à plusieurs reprises. Mais je ne suis pas là pour vendre des illusions.

c'est qu'il y ait un avenir industriel pour le site de GE à Belfort. Il me serait facile de vous dire que l'on va se battre pour les turbines à gaz, mais ce serait mentir aux salariés ! Vous me connaissez suffisamment pour savoir que telle n'est pas ma façon de faire de la politique. En revanche, je suis convaincu qu'il qu'il y a un avenir industriel pour le site de Belfort. Si nous y travaillons tous ensemble, notamment en utilisant les 50 millions d'euros du fonds qui a été mis à disposition pour réindustrialiser ce site avec d'autres projets, il y a de belles perspectives. Il y a des perspectives pour l'aéronautique, qui faisaient partie des propositions que vous m'avez faites et auxquelles je souscris ; nous pouvons y travailler ensemble.

Il y a des perspectives également pour l'hydrogène. Je sais, monsieur le sénateur, que vous soutenez totalement ces projets, et le site de Belfort est très bien placé dans ce domaine. Là aussi, nous pouvons y travailler tous ensemble.

Il faut se battre pour la diversification, vous l'avez dit. Mais il faut aussi se battre pour l'avenir de la France et pour son avenir industriel. Baisser les bras à cause d'une baisse temporaire des commandes de turbines à gaz n'est pas un bon calcul ! Notre indépendance énergétique, notre savoir-faire industriel et nos compétences peuvent être entretenus.

La République En Marche. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur. Hier, dix-huit migrants en provenance du Sri Lanka ont été interpellés par les forces de l'ordre sur une plage de la commune de Bouéni, à Mayotte. Cinq jours plus tôt, c'était un réseau international d'immigration clandestine de migrants en provenance de la République démocratique du Congo qui était identifié et démantelé par le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine, le Gelic, créé spécifiquement à Mayotte en juin 2018. Au lendemain des élections européennes, à l'issue desquelles le Rassemblement national est arrivé largement en tête à Mayotte, une nouvelle filière d'immigration semble faire son apparition dans la commune de Bouéni, qui, je le rappelle, totalise le triste score record de vote pour ce parti, avec 68 % des suffrages. Vous le savez, Mayotte est déjà sclérosée par une immigration clandestine massive en provenance des Comores. Alors même que le plan présenté par Mme la ministre des outre-mer en mai 2018, à la suite du mouvement social contre l'insécurité, produit des résultats tangibles, des kwassas-kwassas accostent encore chaque jour sur nos côtes. sur nos côtes. Monsieur le ministre de l'intérieur, je vous sais déterminé à lutter contre l'immigration clandestine dans ce département. Aussi, pouvez-vous nous détailler l'action du Gouvernement mise en oeuvre à Mayotte pour lutter contre l'arrivée de ces embarcations et, plus généralement, contre l'immigration irrégulière, véritable fonds de commerce du Rassemblement national Comment faire en sorte que les Mahorais cessent de s'en remettre à des partis populistes et extrémistes, qui les oublient sitôt les échéances électorales passées ?

importantes depuis l'Afrique. Là encore, on voit combien ces migrations sont organisées par des gens qui font commerce de la misère humaine et contre lesquels nous devons agir. Il est absolument indispensable

territoriales. Madame la ministre, lors de sa conférence de presse, le 25 avril dernier, le Président de la République a lancé une idée novatrice, en annonçant la création dans chaque canton d'une maison France services où seraient regroupés les services de l'État et tous les opérateurs. Quel ne fut pas mon étonnement Quel ne fut pas mon étonnement ! S'inspirer du modèle canadien, alors que, en France, bon nombre d'élus locaux ont mis en place de telles structures depuis de si nombreuses années ... En effet, depuis la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens avec les administrations, ces maisons France services portent déjà un nom : elles s'appellent les maisons de services au public, les MSAP. Bien auparavant, certaines existaient en tant que relais de services publics. Aujourd'hui, elles sont majoritairement portées par les collectivités, mais également par La Poste.

Je veux bien saluer l'idée affichée de proximité. En revanche, je m'interroge sur l'intérêt de proposer une maison France services dans chaque canton, alors que certains d'entre eux sont parfois plus grands que les communautés de communes. Avons-nous la mémoire si courte que nous en avons oublié que la première de toutes les maisons communes, celle qui appartient à toutes et à tous, qui est connue et reconnue, s'appelle la mairie ? Pendant très longtemps, les services publics dont nous parlonsonttenu des permanences. Peu à peu, celles-ci se sontraréfiées, jusqu'à disparaître. Alors, oui à la proximité, oui à l'accompagnement de nos concitoyens, mais non à des annonces qui masquent la réalité des actions déjà portées et développées par les élus locaux

ou, pour Ariane Chemin, avoir dévoilé qu'un chargé de mission de l'Élysée faisait, à l'occasion, le coup de poing lors de manifestations, et qu'il entretenait des relations pour le moins douteuses. Ces convocations, cette volonté d'intimidation, s'inscrivent dans un contexte plus large de défiance du Gouvernement vis-à-vis de ce contre-pouvoir qu'est la presse. Je pense notamment à l'arrestation de Gaspard Glanz lors de la manifestation du 1 mai

Face à ce climat inquiétant et à ce qui s'apparente à une volonté d'intimider les journalistes, notre groupe tient à rappeler son attachement aux libertés fondamentales, à la liberté de la presse et à la protection des sources, sans lesquelles l'information ne serait plus la même. À l'inverse, le Gouvernement et le Président de la République continuent de justifier, sous couvert de sécurité nationale ou de secret défense, l'injustifiable. Car comment appeler autrement la convocation de journalistes et du patron du groupe par un service censé lutter contre les menaces terroristes ? de la justice, quand le Gouvernement va-t-il mettre un terme à ces pratiques qui fragilisent la liberté de la presse et ternissent considérablement l'image de liberté de notre pays à l'international ?

Laissez-moi tout d'abord vous dire, madame Claudine Lepage, que, tout comme vous, le Gouvernement est attaché à la liberté d'informer et à la protection du secret des sources. Mais nous devons également protéger les agents qui concourent à la sécurité de notre pays. Concernant les affaires évoquées, je vous rappelle que, en tant que garde des sceaux,

qui est de la convocation de Mme Ariane Chemin, journaliste au, celle-ci est intervenue dans le cadre d'une enquête préliminaire qui est placée, vous le savez, sous le contrôle du procureur de la République de Paris. a été ouverte à la suite du dépôt de plainte d'un membre des forces spéciales dont l'identité avait été révélée par ce journal. S'agissant de la convocation par la DGSI d'un journaliste du média que vous avez évoquée, elle intervient, là encore, dans le cadre d'une procédure judiciaire menée sous l'autorité d'un magistrat. Cette enquête préliminaire a été confiée à la DGSI par le procureur de la République de Paris, du chef de compromission du secret de la défense nationale. Juridiquement, ces éléments sont potentiellement constitutifs d'une infraction pénale. Je rappelle que, dans le cadre d'une audition libre comme d'une garde à vue, les personnes convoquées disposent de droits, et en premier lieu de celui d'être assisté d'un avocat pendant leur audition. Je rappelle également qu'une telle convocation ne préjuge en rien l'éventualité de poursuites qui pourraient être diligentées à l'encontre de ces journalistes. Enfin, il appartiendra au seul procureur de la République de juger des suites à donner. Cette convocation, madame la sénatrice, ne doit en aucun cas être lue comme une tentative d'intimidation ou de menace. Non, bien sûr ! Je vous redis ici qu'elle est intervenue dans un cadre juridique précis, respectueux de l'État de droit, et que, tout comme vous et l'ensemble des sénateurs, le Gouvernement est particulièrement attaché à la liberté de la presse.

Monsieur le ministre, ce changement n'a l'agrément ni des communes forestières ni de leurs fédérations. Plusieurs milliers de délibérations ont d'ailleurs été prises pour protester

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande du débat dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mis en place au milieu des années quatre-vingt, le bac professionnel souffre depuis l'origine d'un déficit d'identification, puisqu'il a été créé autant pour répondre à une nécessaire professionnalisation en France que pour atteindre le très contestable objectif des 80 % d'une classe d'âge au niveau du bac. L'article L. 335-1 du code de l'éducation nationale dispose que l'enseignement technologique et professionnel « contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification et qu'il « doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures ». Force est de constater que la réforme conduite actuellement par votre ministère laisse perplexes bon nombre de professeurs de lycée quant à la réalisation de ces objectifs. suite de plusieurs interpellations de ces professeurs, syndiqués ou non, et au regard de la faible visibilité de cette réforme dans le débat public et dans les médias, le groupe Les Républicains a souhaité que l'ensemble des sénateurs puisse vous entendre, monsieur le ministre, répondre aux multiples questions qui émanent du terrain. Je me félicite évidemment de la tenue de ce débat, mais je conviens que la tâche n'est pas facile, puisqu'il nous faut interpeller sans caricaturer, définir sans enfermer et finalement dire sans stigmatiser. Tout d'abord, il est essentiel de rappeler qu'un lycéen sur trois est inscrit dans la voie professionnelle. C'est considérable, et la réussite de ces jeunes est un enjeu national. Mais comment concilier dans une même formation un objectif d'insertion professionnelle immédiate avec un objectif de facilitation de la poursuite d'études ? Claude Lelièvre, historien de l'éducation, reconnaît même que « personne, depuis Chevènement, n'a été capable de dire ce que devait être l'enseignement professionnel

Dans la filière gestion-administration, par exemple, qui est la plus importante de la voie professionnelle, seuls 34 % des jeunes diplômés sont en emploi sept mois après l'obtention de leur baccalauréat. Quant à la poursuite d'études, le BTS reste la voie « royale » pour ces bacheliers. Mais, là encore, le taux de réussite n'est pas satisfaisant : les bacheliers professionnels accusent un écart de 20 points sur les bacheliers technologiques et de plus de 30 points sur les bacheliers généraux. Une réorganisation de la voie professionnelle, dans le cadre de la réforme plus globale du baccalauréat, est donc, sur le papier, une bonne idée. Les acteurs du lycée pro y étaient d'ailleurs favorables. Sur le papier, justement, la réforme que vous avez engagée peut paraître séduisante sur plusieurs points. J'en ai noté deux : tout d'abord, la création des campus d'excellence a pour ambition de conférer une meilleure visibilité, même si elle risque de renforcer les disparités et de créer une mise en concurrence entre les établissements l'accent mis sur les formations de pointe aux métiers d'avenir contribue à une nécessaire modernisation des filières. Cependant, si on laisse de côté les formules de communication bien huilées, le détail des mesures est plus nuancé. Instaurer la classe de seconde par famille de métiers tend à reculer le choix de l'orientation à la fin de la seconde et non de la troisième. Chacun sait, et ce n'est pas propre à cette génération, que ce choix est difficile pour des jeunes de 14 ans ou 15 ans et pour leur famille. confrontés le plus souvent à un échec scolaire qui les enferme en réalité dans un choix par défaut. Mais cette mesure comporte un risque de « dé-spécialisation » des jeunes et, en toute logique, devrait conduire à un allongement du temps de formation professionnelle. Il n'en est rien dans la réforme proposée, qui, au contraire, réduit le nombre d'heures d'enseignement. Nous en venons à la mesure qui inquiète le plus le corps enseignant et sur laquelle la représentation nationale a été le plus alertée : la perte de quatre heures par semaine d'enseignement général. Sans caricature ni stigmatisation, partons d'abord d'un constat : les jeunes lycéens professionnels sont issus de milieux les plus fragilisés socialement, financièrement et culturellement. S'ils se destinent à une formation très professionnalisante, ils ont le plus grand besoin d'un enseignement dans des matières comme le français, l'histoire-géographie ou l'éducation civique et morale. ! Pourtant, ces trois matières combinées ne feront bientôt plus l'objet que de deux heures de cours par semaine, ce qui est évidemment très insuffisant pour former des citoyens éclairés, conformément à l'objectif que vous vous êtes fixé, monsieur le ministre. Même si la réforme permet la co-intervention des professeurs, qui est d'ailleurs déjà mise en place dans les faits dans beaucoup de lycées, le français qui sera enseigné en atelier, par exemple, ne sera qu'un français dit « utilitaire ». les enseignants exerçant en lycées professionnels ne peuvent être assimilés à des formateurs en recrutement. Cette réduction horaire pénalisera l'ensemble des élèves, quel que soit leur choix à l'issue du baccalauréat. S'ils visent une insertion professionnelle, des jeunes qui ne maîtrisent pas correctement notre langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, auront plus de difficultés à entrer sur le marché du travail. S'ils s'inscrivent dans une poursuite d'études, ils souffriront encore davantage de lacunes en français ou en mathématiques, déjà largement constatées dans des filières comme les DUT ou les BTS. que l'on ne me parle surtout pas de l'élargissement du dispositif d'accompagnement personnalisé, véritable « tarte à la crème » des réformes de l'éducation nationale depuis vingt ans, qui ne repose sur aucun programme, dont l'application varie d'un professeur à l'autre, et dont on attend de constater l'inutilité pour pouvoir supprimer ultérieurement de nouvelles heures ! Le fort absentéisme révèle d'ailleurs à lui seul tout l'intérêt que les élèves Un autre pan de la réforme prévoit la mixité des publics et des parcours, avec la généralisation de l'apprentissage. Nous l'avons assez répété sur ces travées, l'apprentissage est pour nous une composante essentielle de la formation des jeunes, et tout ce qui permet de l'encourager est une bonne chose. il nous faut être vigilants quant à sa réalisation concrète. Comment, en effet, concilier les absences prolongées de certains avec le continuum des cours des autres ? De plus, en dehors de toute stigmatisation, nous savons que les jeunes inscrits dans la voie professionnelle n'ont pas toujours tous les codes : trouver un contrat d'apprentissage peut parfois se révéler pour eux un vrai casse-tête.

Monsieur le ministre, pour présenter votre réforme, vous parlez de la voie professionnelle comme d'une « nouvelle voie vers l'excellence ». Force est de constater que bon nombre d'acteurs de l'enseignement professionnel doutent des capacités de vos mesures à répondre à cet objectif. À mon sens, contrairement à l'ambition affichée au départ, cette réforme ne conduira pas à ne plus considérer cette filière comme une voie « de garage », dans laquelle on envoie les collégiens qui rencontrent le plus de difficultés. Elle ne permet pas de combattre le sentiment, constaté chez la majorité des jeunes qui arrivent en seconde professionnelle, de dévalorisation, de démotivation, voire de pessimisme quant à leur avenir. elle ne fait nullement écho à l'abattement des professeurs, tellement désabusés qu'ils renoncent à engager un mouvement de protestation et font massivement des demandes de mutation. Bien sûr, les textes réglementaires ont presque tous été pris, et les lycées sont d'ores et déjà en train de s'organiser, parfois dans l'urgence, pour les mettre en oeuvre dès la rentrée prochaine. Notre débat n'a donc pas pour ambition de modifier votre trajectoire, mais il a le mérite d'engager une réflexion qui devra porter sur le long terme.

En la tenant pour une priorité essentielle, je veux signifier que l'enseignement professionnel n'est pas marginal dans notre système et n'est pas la dernière de nos préoccupations. Il est au contraire au coeur de notre volonté de progrès, non seulement en raison de l'enjeu social que vous avez rappelé, mais aussi parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Il s'agit non pas seulement d'améliorer grandement le parcours d'élèves socialement défavorisés et constituant une partie des décrocheurs scolaires de notre pays, mais aussi de préparer aux métiers du futur ceux qui suivent ce parcours.

formule trouvera une incarnation au cours des prochaines semaines lorsque nous présenterons les premiers projets de campus conçus avec des régions. Nous partirons de lycées professionnels existants ou parfois de projet,

auront envie d'aller dès la fin de la troisième, non parce qu'ils ont un mauvais bulletin scolaire, mais parce qu'ils ont envie d'apprendre autrement et de se diriger vers des métiers d'avenir. Le fonctionnement en campus va de pair avec le fonctionnement en réseau. Tout lycée professionnel de France, dans le futur, se trouvera désormais à la fois dans un réseau géographique et dans un réseau thématique.

est d'offrir un panel de possibilités à chaque élève de France voulant s'inscrire en lycée professionnel. C'est le sens du fonctionnement en réseaux géographiques. Nous voulons aussi des réseaux thématiques

Nous sommes dans une logique de formation tout au long de la vie. Et c'est cette logique qui a un impact en amont sur ce qu'est le lycée professionnel. Notre ambition, je vous l'accorde, monsieur le sénateur, est très forte,

Je pense à l'esprit d'équipe. Je pense aussi à l'instauration d'une pédagogie d'équipe et de projets, qui sont des compétences fondamentales dans la vie professionnelle et qui pourront avoir un impact sur des modalités pédagogiques en dehors de l'enseignement professionnel.

que suit un élève n'est certainement pas un indicateur de bon fonctionnement d'un système. Si tel était le cas, le lycéen professionnel français serait aujourd'hui le meilleur lycéen du monde, car il bénéficie de 34 heures à 35 heures de cours hebdomadaires. Or il décroche, il ne suit pas, il assiste à des cours d'enseignement général dans des classes de 35 élèves. Soit on fait semblant d'ignorer ces réalités et on formule des critiques assez faciles. Soit on les prend à bras-le-corps, en s'appuyant sur les pratiques pédagogiques qui fonctionnent. C'est ce que j'ai fait,

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel vient considérablement modifier le financement les CFA. À la suite des premiers retours des coûts contrats en apprentissage, les coûts pour certaines formations seront inférieurs aux coûts régionaux. Par exemple, en Vendée,

Si ces différences étaient confirmées sur tous les établissements ayant un cycle de formation CAP, brevet professionnel ou bac pro, cela représenterait un manque à gagner de plus de 100 000 euros. Par ailleurs, dans les coûts, la question du financement des investissements reste en suspens. Avant la réforme de 2018, les investissements pouvaient être financés par la région, car l'apprentissage était de la compétence de cette dernière. À l'heure actuelle, nous ignorons si c'est avec le coût contrat que les établissements CFA devront financer les investissements et s'ils auront, notamment, la capacité de poursuivre ces investissements pour adapter les plateaux techniques. Aujourd'hui, les textes annoncent des financements complémentaires aux coûts contrats pour accompagner l'hébergement, la restauration et l'aide au premier équipement, ainsi que pour aider à la mobilité internationale. Mais, à ce jour, le flou demeure et les établissements professionnels sont contraints

Que deviendront ces jeunes, sachant que,, les classes de « troisième prépa métiers » ont été ouvertes, mais pas dans les CFA ? Au vu de ces éléments, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous éclairer sur la façon dont seront déterminés les coûts, sur les modalités d'attribution des financements complémentaires et, enfin, sur le devenir des jeunes, qui ne peuvent plus bénéficier du DIMA au sein des CFA ? La parole

à la suite des propos de M. le sénateur Piednoir. Il est en effet important de rappeler que la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel a ouvert une nouvelle phase de l'apprentissage, une nouvelle étape, à laquelle l'enseignement professionnel contribue.

en voie générale, en voie technologique, en voie professionnelle ou en apprentissage, et cela a eu un impact. Comme vous l'avez rappelé, la responsabilité de définir le montant du coût du contrat d'apprentissage appartient désormais aux branches professionnelles. Il s'agit d'un coût national : chaque diplôme ou titre aura un coût précis, qui s'appliquera uniformément sur l'ensemble du territoire.

déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, ou encore du premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation, selon les besoins définis par domaine d'activité, identiques pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, avec un plafond de 500 euros. Les frais de mobilité

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, connaissez-vous celles et ceux que l'on appelle les « nouveaux artisans » ? Ils sont boulangers, coiffeurs, restaurateurs ou encore agriculteurs et ils ont décidé de se reconvertir volontairement pour répondre, enfin, à leur volonté d'exercer un métier manuel. Ils abandonnent parfois des carrières prestigieuses pour retourner sur les bancs de l'école et apprendre un nouveau métier, celui dont ils rêvaient vraiment. Ces jeunes en quête de sens et de concret forcent l'admiration. Ils dénoncent aussi, en creux, le mal profond qui ronge l'enseignement professionnel. Parce qu'il n'a pas été suffisamment encouragé et valorisé par les pouvoirs publics, celui-ci est trop souvent perçu comme une voie de garage. Des décennies de politiques malheureuses ont ainsi organisé un immense gâchis, en remplissant des filières d'élèves condamnés à des parcours scolaires et professionnels de second rang. En effet, l'enseignement professionnel est encore trop souvent la dernière option envisagée. Pourtant, l'enseignement professionnel semble la pièce manquante du puzzle, dans un pays où plus d'un jeune sur cinq est encore au chômage. À l'heure où nous cherchons à diffuser plus largement l'envie d'entreprendre, cette voie pourrait bien constituer l'un des leviers pour redynamiser notre économie et réconcilier notre société avec elle-même. Monsieur le ministre, comment comptez-vous lutter contre le blocage culturel qui plombe cette filière ? Comment valoriser efficacement la voie professionnelle auprès des jeunes et des familles ? La parole est à M. le ministre. Monsieur le sénateur, votre

Estrosi Sassone. Monsieur le ministre, les lycées d'enseignement général, technologique et professionnel ainsi que les CFA partagent la même ambition, quelle que soit l'orientation choisie par les élèves

% en lycée professionnel -met en péril la possibilité pour les élèves d'accéder aux filières supérieures de BTS, faute d'une formation suffisante au regard des exigences. Ce constat est unanimement partagé par les professeurs, qui signalent également que les nouvelles heures d'enseignement en co-intervention réduisent les mathématiques, le français et les enseignements

de la nouvelle répartition de la taxe d'apprentissage va engendrer des inégalités, alors que cette taxe a pour objet de favoriser l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire. La perte de redevance pour la tranche « hors quota » est une inquiétude légitime des enseignants, car ce solde, réduit de 23 % à 13 %, est destiné aux formations professionnalisantes en lycées professionnels. Monsieur le ministre, comment comment compenser cette perte de moyens tout en garantissant la qualité et l'attractivité de ces filières, qui ont besoin d'équipements ? Par ailleurs, comment comptez-vous former de futurs professionnels accomplis, passionnés et motivés, alors que le volume horaire d'enseignement ne cesse de baisser ?

pour certains types d'enseignement. Les professeurs sont malheureux de cette situation, les conditions générales ne permettant pas l'attractivité de l'enseignement professionnel. La co-intervention, pour laquelle nous ne

comme les séjours professionnels, les visites d'entreprises ou les visites de sites européens sont financés sur la redevance « hors quota ». Demain, ces projets pourraient être purement et

Mme Françoise Cartron. Monsieur le ministre, quarante-huit heures après un rendez-vous électoral européen majeur, je souhaitais aborder aujourd'hui la possible montée en puissance du programme Erasmus+ à destination des apprentis et des lycéens professionnels. Le 23 mai dernier, vous avez dévoilé, dans un quotidien national, un nouveau système d'équivalence, afin de conduire plus de la moitié des futurs professeurs, notamment dans l'enseignement professionnel, à faire un stage ou un séjour dans un autre pays d'Europe. De même, les élèves de CAP ou de bac pro pourront obtenir des points en plus s'ils effectuent une mobilité. L'objectif d'encourager les mobilités européennes et de les valoriser afin de les rendre plus accessibles à des jeunes, en particulier ceux qui sont issus de milieux modestes. Vous appelez à un « Bologne de l'enseignement professionnel », avec des équivalences par-delà les frontières, qui contribuerait à créer un espace européen de l'enseignement supérieur. Nous le savons, cet espace ne sera viable que s'il ne laisse aucun territoire de côté. Monsieur le ministre, quels sont les objectifs en la matière, en nombre de bourses, en dispositifs d'accompagnement ? Combien d'élèves de l'enseignement professionnel pourraient être concernés ? Quelle action est-elle possible au niveau européen ? Je pense également à la possibilité d'un parrainage ou marrainage de la part des étudiants étrangers en mobilité en France et de la part des étudiants français revenus de leur mobilité. effet, derrière la possibilité matérielle d'une mobilité, il y a aussi le désir de celle-ci, qu'il est possible de susciter en faisant tomber certaines barrières symboliques auprès des élèves les plus éloignés,

Nous pouvons donc doubler le nombre de mobilités d'ici à trois ans, pour atteindre 40 000 lycéens et apprentis concernés et 20 000 jeunes passant l'épreuve de mobilité, laquelle est

de « mener une analyse approfondie concernant la situation de l'affectation des bacheliers technologiques et professionnels dans l'enseignement supérieur et

Parcoursup, le nombre de réponses favorables pour les lycéens issus des filières professionnelles était nettement moindre. Et les premiers chiffres disponibles montrent que, malheureusement, pour l'épisode 2 de Parcoursup, c'est exactement la même chose. Les discriminations

en dépit de l'excellence des formations, force est de constater que le taux d'échec demeure important dans l'enseignement professionnel. Malgré vos propos très positifs, auxquels on ne peut que souscrire,

le lycée professionnel est celui qui coûte le plus cher, a le plus d'heures de cours et n'est pas synonyme de réussite ». Est-ce dans la continuité de ce raisonnement que vous réduisez le volume d'heures d'enseignement global à 30 heures par semaine, notamment celui des matières générales Le contenu des programmes lui-même a été pour le moins resserré ! Ces aspects risquent fort de minorer la qualité du bac pro et, par là même, l'insertion professionnelle des bacheliers. En classe de seconde, vous avez annoncé la création des « familles de métiers ». Leur mise en oeuvre effective apparaît toutefois difficile dans certains territoires. Comment cette mesure sera-t-elle appliquée dans les académies qui ne disposent pas de tous les bacs d'une même famille de métiers ? Cette première année, très généraliste, aura également pour conséquence de déprofessionnaliser les bacheliers professionnels, ramenant le bac pro à deux années de préparation réelle seulement, alors que les entreprises expriment avec force leur besoin de main-d'oeuvre spécialisée. Le Conseil supérieur de l'emploi, de décembre dernier. Monsieur le ministre, il apparaît que votre réforme ne déploie pas des moyens à la hauteur des enjeux de l'enseignement professionnel, qui contribue pourtant

Madame la sénatrice, la question que vous posez est importante. J'y ai répondu s'agissant des critères de gestion et, encore une fois,

pour le bac général et technologique, où nous fixons des horizons de grands domaines, et non de métiers précis. Pour la rentrée de 2019, nous commençons par trois familles : métiers de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics, métiers de la relation client et métiers de la gestion administrative, du transport

des élèves choisissant cette voie. En effet, le français, l'histoire-géographie et l'éducation morale et civique perdent un volume total de 113 heures sur trois Or cet enseignement général est indispensable à la formation de ces jeunes élèves, au parcours parfois chaotique et pour qui le lycée professionnel est souvent la seule chance d'avoir un emploi ou de poursuivre des études supérieures. Aujourd'hui, 38 % des élèves de lycées professionnels poursuivent leur cursus après le bac. Ils n'étaient que 17 % en 2000. C'est une belle progression ! Toutefois, leurs résultats en BTS sont mitigés : seuls 62 % d'entre eux décrochent le diplôme, pour 87 % des bacheliers généraux. En réduisant la part de l'enseignement disciplinaire, on risque de creuser l'écart entre le lycée professionnel et la poursuite d'études. Les lycéens professionnels ne doivent pas être privés de culture générale. C'est une erreur de croire qu'ils n'en auront pas besoin. Privilégier la pratique et la technique est certes une bonne chose, mais cela ne doit pas se faire au détriment de matières fondamentales pour le développement intellectuel de ces élèves. Seul un socle de valeurs culturelles et citoyennes permettra à ces jeunes de s'adapter aux évolutions du monde et aux métiers qu'ils pratiqueront. Monsieur le ministre, comment comptez-vous pallier la baisse de ce nombre d'heures d'enseignement des matières générales en lycée professionnel ? La parole est à M. le ministre. Madame la sénatrice,

de nombreux élèves en échec scolaire au collège retrouvent confiance et réussite au lycée professionnel. Un enseignement avec des pratiques pédagogiques souvent très innovantes, dont l'enseignement général s'inspire

-rénové le statut des apprentis en s'attachant à corriger son opacité et sa complexité, ainsi qu'à effacer les travers qui contribuaient à en donner une image largement dégradée. Or l'augmentation de la rémunération des apprentis, le remplacement du système d'aides par une aide unique aux employeurs d'apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés et la suppression des exonérations totales de charges sociales se traduisent par un surcroît significatif pour les employeurs dans certaines situations ; cela concerne particulièrement les apprentis plus âgés. Par ailleurs, l'aide unique aux employeurs d'apprentis ne couvre pas les diplômes et titres de niveau Or, si cette réforme a, en principe, pour objectif d'améliorer largement le dispositif, il ne faut pas qu'elle induise des conséquences financières délétères pour les employeurs, ce qui les découragerait. Par exemple, le coût global d'un apprenti de 27 ans embauché dans une entreprise de moins de 250 salariés pour préparer un CAP boulanger,

Ce delta a été constaté dans d'autres secteurs comme la coiffure. Compromis entre productivité et observation, l'apprentissage d'un jeune représente, malgré tous ces avantages, une charge pour l'entreprise, qu'il ne faut pas négliger. Aussi, je souhaiterais recueillir votre avis sur deux points d'amélioration, monsieur le ministre. d'une éventuelle révision du système de rémunération des apprentis, à savoir la création d'un salaire minimum légal de l'apprenti basé sur le seul critère du niveau de

Développer l'apprentissage implique, entre autres, de simplifier les démarches des employeurs afin d'augmenter le nombre de contrats offerts aux jeunes. Désormais, dans les entreprises de moins de 250 salariés lorsqu'est signé un contrat d'apprentissage pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au

dès que le contrat d'apprentissage est enregistré par la chambre consulaire, l'aide est versée par l'Agence de services et de paiement chaque mois par anticipation de la rémunération. Le montant de l'aide unique est dégressif : 4 125 euros au maximum pour la première année d'exécution du contrat ; 2 000 euros au maximum pour la deuxième année et 1 200 euros pour la troisième. Un simulateur de calcul de rémunération est disponible sur le portail de l'alternance. Par exemple, s'agissant d'un apprenti de 16 ans qui prépare un CAP dans une entreprise de moins de onze salariés, le reste à charge mensuel pour l'employeur, déduction faite de l'aide unique et des exonérations de cotisations sociales, s'élève à 73 euros par mois la première année et à 436 euros la seconde année. Par ailleurs, vous avez insisté sur l'apprentissage après le baccalauréat. C'est un point fort de la France, vous le savez, et, là aussi, des moyens publics viennent en appui des employeurs.

Ainsi, d'après cette étude, un jeune sur deux déclare ne pas avoir été bien accompagné dans son établissement pour ce qui concerne son projet d'orientation et un jeune sur cinq estime qu'il n'a pas eu le choix de son orientation.

La voie générale est souvent plébiscitée par le corps professoral et les professionnels de l'orientation. Pourtant, nombre de bacheliers échouent ensuite à l'université ou se lancent dans des études parfois longues et se rendent compte, en cours de route, qu'ils ne parviendront pas à les finir ou qu'ils se sont trompés de voie.

pourriez-vous nous préciser les mesures que le Gouvernement entend mettre en place pour faire en sorte que l'enseignement professionnel retrouve ses lettres de noblesse et redevienne le pourvoyeur de jeunes employés formés pour les filières professionnelles qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être, et ce en adéquation avec le marché de l'emploi ? Deuxièmement, ne pensez-vous pas que la professionnalisation des parcours devrait être abordée dès le collège, à partir de 14 ans, afin d'éviter le décrochage scolaire de certains jeunes, qui sont confrontés à des notions parfois trop abstraites dans les formations classiques ?

en matière d'orientation. Concrètement, cela signifie que, désormais, les régions ont un rôle direct pour ce qui concerne les heures d'orientation que nous dédions aux différentes classes du collège et du lycée.

déspécialisation et déqualification par la réduction des 80 formations existantes à quelques familles de métiers ; diminution des heures de cours ; personnalisation à outrance des parcours ; suppressions de postes d'enseignants ; nombre d'élèves par classe

« Arts de la reliure et de la dorure ». Là-bas, comme ailleurs, cette réforme suscite de légitimes inquiétudes. En effet, la baisse de la part de l'enseignement général dans les formations est considérée comme paradoxale par rapport, je le répète, à l'ambition d'« excellence » affichée. Si je reconnais que l'école, en particulier l'enseignement professionnel, a pour rôle de préparer des jeunes au monde du travail, je n'oublie pas qu'elle doit aussi, et surtout, former des citoyens et des citoyennes. Or les élèves seront privés chaque semaine de plusieurs heures de français, de mathématiques, d'histoire-géographie, et l'enseignement de ces matières générales sera principalement au service du métier et des seules compétences techniques. Très souvent, Très souvent, nous le savons, l'enseignement professionnel permet à des jeunes qui se sentaient exclus du savoir et de la réussite scolaire de se remettre sur les rails. L'équilibre entre des disciplines professionnelles destinées à l'apprentissage d'un métier et des matières générales qui ne sont pas systématiquement connectées à la profession est essentiel. cette réforme appauvrit les contenus des formations et risque de priver les élèves d'une insertion professionnelle véritablement qualifiante, comme de la possibilité de poursuivre des études. Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi le fait de réduire les enseignements généraux dans la formation professionnelle des élèves permettra à ces derniers d'accéder à « l'excellence »

personnalisation à outrance ». Je ne sais pas ce que peut être la personnalisation à outrance, mais plus on personnalise, mieux c'est ! Il est évidemment nécessaire d'avoir une approche personnalisée du parcours de l'élève.

Bories. Madame la présidente, monsieur le ministre, de nombreux professionnels de tous horizons de mon département font remonter du terrain une pénurie croissante de personnes correctement formées aux besoins de l'entreprise. Pourtant, l'enseignement professionnel représente plus de 200 CAP et 100 bacs professionnels différents. Par ailleurs, dans mon territoire du Gard rhodanien, situé en limite géographique départementale et régionale, la plupart des formations professionnelles situées à moins de vingt kilomètres sont installées dans la région voisine, avec un réseau de transport en commun accessible.

permettre enfin à ces jeunes d'accéder à ces lycées professionnels en se fondant sur un raisonnement de bassin économique et d'infrastructures de transport en commun et non plus sur les limites d'académie ? propos en préambule, porte sur l'adéquation entre les demandes de formation et les besoins actuels des entreprises, notamment dans leur secteur géographique. Certaines entreprises n'hésitent plus à ouvrir leur propre centre de formation.

le littoral français est le deuxième le plus étendu au monde. Il est une chance pour notre pays et un levier de croissance à ne pas négliger. À Marseille, avec près de soixante kilomètres de façade maritime, la ville dispose d'importants atouts dans ce domaine et pourrait même à l'avenir être à l'avenir être une vitrine pour notre pays. Pour ce faire, il est primordial d'encourager nos jeunes à se tourner vers les métiers de la mer, en créant un pôle des métiers d'activités maritimes. Au-delà des traditionnelles activités portuaires, des filières émergentes, comme la protection de l'environnement et l'aménagement du littoral, l'exploitation des ressources biologiques marines, les énergies marines renouvelables ou encore la promotion de la culture de la mer, sont autant d'activités porteuses à stimuler. Dans une ville où le chômage frappe plus qu'ailleurs et où de nombreux jeunes souhaitent rapidement s'orienter vers un parcours scolaire professionnalisant, ces activités représentent une chance, voire une aubaine.

Comme vous le savez, les Segpa ont été créées en 1996, afin de répondre aux difficultés rencontrées par les élèves en situation d'échec scolaire important. Ces classes, restreintes en nombre d'élèves, ont pour vocation de mener les élèves vers une qualification diplômante, le plus souvent dans une filière d'enseignement professionnel.

que les formations préparant à ces professions bénéficient d'une image positive et attractive. Or, si l'on cantonne les enseignements manuels et la préparation au lycée professionnel aux seuls élèves en difficulté, on associe indirectement la profession manuelle à l'échec scolaire.

où l'enseignement général et l'enseignement professionnel pourraient cohabiter de manière constructive, afin de les accompagner vers les filières professionnelles, tout en ne négligeant pas l'acquisition des savoirs fondamentaux.

: nous renforçons les différentes dimensions de l'école inclusive, donc aussi du collège inclusif. Vous le savez- c'est l'une des caractéristiques de la rentrée prochaine -, plus les Segpa sont justifiées dans leurs particularités,

Fournier, pour une meilleure articulation entre la scolarité, l'orientation professionnelle et l'accompagnement de proximité des jeunes, qu'ils soient élèves, étudiants ou apprentis, dans leur parcours de formation, en insistant sur l'objectif de déboucher sur un métier porteur d'avenir. Le travail porté sur la question de l'apprentissage en France vaut pour l'enseignement professionnel. Nous n'avons pas là deux entités qui s'affrontent, puisque l'objectif est commun : la réussite des jeunes, des jeunes, laquelle passe par un encadrement et une animation du système éducatif professionnel à la hauteur des besoins des métiers et des jeunes. Je voudrais dire à cette occasion, comme je l'ai fait lors de l'examen de la loi de 2018, que l'État, par l'intermédiaire de l'éducation nationale, ne doit pas se priver de la connaissance les régions, mais favoriser les pratiques de formation en alternance. L'enseignement professionnel ne doit plus être un choix par défaut. Il concerne un quart des lycéens, et il n'est pas le parent pauvre de l'enseignement général ou de l'apprentissage. Les campus de formation professionnelle existent déjà. Vous avez bien raison de vouloir les généraliser. Par exemple, dans les métiers de la restauration, les métiers de bouche et de l'hôtellerie, à Dardilly, près de Lyon, le lycée Rabelais, qui comprend aussi un CFA, fonctionne en relation avec la filière gastronomique de la région lyonnaise et porte des projets européens. Cependant, dans votre volonté affirmée de sonner la mobilisation générale, il nous semble aberrant, monsieur le ministre, que la compétence des régions ait été réduite à une simple information sur l'orientation.

Je tiens à votre disposition à la fois la convention signée ce matin et le dossier qui l'accompagnait, lequel permet de voir que les régions se sont déjà préparées pour cela. Elles se sont préparées notamment pour occuper ce domaine horaire que nous avons défini pour chaque année d'enseignement. C'est important

pour l'éducation -, mais à un véritable partenariat entre les régions, l'État et l'éducation nationale. Cela signifie aussi que les régions

réplique. Monsieur le ministre, je vous ai posé cette question, car, vu ce qui s'est passé ce matin, je comprends encore moins que vous n'ayez pas accepté les propositions du Sénat

voire de les contraindre à fermer leurs portes. La région d'Île-de-France est alertée, mais je souhaite surtout que l'État ne se désintéresse pas trop vite d'un CFA qui est vraiment la référence des métiers d'art en France.

puisque ce projet, porté par Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants, le GNI de l'hôtellerie-restauration, a pour ambition d'implanter à Paris la grande école hôtelière gratuite qui lui fait défaut. Un établissement pour les professionnels, géré par les professionnels, qui pourra rivaliser avec les plus grandes références internationales, et où 1 1 200 apprenants seront formés à plus de 25 métiers de l'hôtellerie-restauration, avec notamment un hôtel d'application, ce qui n'existe pas à Paris.

formations pour tout jeune de 16 ans à 18 ans quand celui-ci n'est pas déjà dans une formation ou dans un emploi. Elle crée donc aussi un contexte très favorable pour ce type d'initiative. Nous allons donc voir émerger, au cours des prochains mois et des prochaines années, de grands campus, qui correspondent aux grands domaines d'embauche.

au service des jeunes. Je pense que nous aurons ainsi un modèle français de formation professionnelle extrêmement intéressant. Nous nous serons inspirés en partie de nos voisins, comme la Suisse et l'Allemagne, que nous avons beaucoup étudiés, mais il y en a eu aussi d'autres, tout en faisant quelque chose de proprement français, parce que notre tradition d'enseignement scolaire professionnel est magnifique. Elle constitue un atout considérable.

Dumas, pour la réplique. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je voulais vraiment attirer votre attention sur ces métiers et ces secteurs, qui touchent à la tradition, à l'excellence française et à la transmission du savoir-vivre français dans le monde.

qui entrera en vigueur à la rentrée de 2019. Je voudrais, en conclusion de ce débat, remercier tous nos collègues qui sont intervenus pour relayer les inquiétudes des élèves, des parents et du corps enseignant. Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une réflexion articulée autour des réformes du baccalauréat, de l'accès aux études supérieures, de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Il faut savoir est en voie professionnelle. L'enseignement professionnel, ce sont aujourd'hui 665 000 élèves scolarisés et plus de 300 spécialités, même si, en réalité, trois spécialités dans le secteur des services accueillent à elles seules les deux tiers des élèves gestion-administration ; commerce ; accompagnement, soins et services à la personne. Voilà tout juste un an, le 28 mai 2018, vous aviez présenté, monsieur le ministre, vos propositions pour un lycée professionnel transformé, qui formerait les talents aux métiers de demain. Fort du constat que la filière professionnelle connaissait de très belles réussites, vous aviez alors souligné les difficultés dont souffrait la voie professionnelle : un déficit d'attractivité lié à une valorisation insuffisante des formations professionnelles ; une offre de formation pas toujours adaptée aux besoins des territoires et aux enjeux d'avenir ou encore des taux d'insertion insuffisants. Ainsi, quelque 51 % des titulaires d'un CAP et 34 % des bacheliers professionnels étaient au chômage sept mois après l'obtention de leur diplôme. Nous ne pouvions alors que partager ce constat et saluer l'ambition d'une réforme qui visait à remédier aux déséquilibres de l'enseignement professionnel et à améliorer sa lisibilité pour les élèves et leurs familles. Sur les neuf leviers du rapport Calvez-Marcon du 22 février 2018 sur la voie professionnelle scolaire, trois ont été retenus : des campus de nouvelle génération, dits « d'excellence », censés incarner une offre de formation riche, claire et attractive des formations de pointe en phase avec les grands enjeux du XXI siècle ; des parcours éclairés par une pédagogie innovante, moteur de réussite. En d'autres termes, il s'agit de relier les enseignements généraux et professionnels pour donner plus de sens. Il est essentiel de le rappeler, l'objectif du lycée professionnel, c'est de proposer un enseignement en alternance avec l'entreprise et ses métiers, afin de faire acquérir des compétences et des connaissances générales et professionnelles, dans divers secteurs et à différents niveaux de formation. L'enseignement dispensé a deux finalités : l'insertion professionnelle, certes, mais aussi la poursuite des études. Or, sur ce dernier point, la mise en oeuvre de la réforme pose des questions et inquiète. Le ministère annonce de nouvelles grilles horaires et une nouvelle organisation des études. Les périodes de formation en milieu professionnel sont revues à la baisse, les 22 semaines en vigueur devenant un maximum. L'horaire hebdomadaire est également réduit, au détriment de l'enseignement général. Le français, l'histoire-géographie et l'éducation morale et civique, qui forment une seule discipline, vont perdre 113 heures sur trois ans, sans compensation par la co-intervention. À cela s'ajoute encore la baisse des enseignements en langues, qui passent de 349 heures à 265 heures, en contradiction avec le souhait de développer Erasmus. Quelles conséquences auront ces baisses sur les projets des élèves ? Aujourd'hui, sur les 100 000 élèves des lycées professionnels qui poursuivent leurs études après le bac, 37 000 seulement sont admis en BTS. Or seuls 62 % de ces élèves décrochent leur diplôme, contre 87 % pour les bacheliers généraux. Ne va-t-on pas creuser encore plus le fossé entre bacheliers professionnels et bacheliers généraux ? Si la réforme avait pour but d'améliorer la lisibilité de l'enseignement professionnel et visait l'excellence, le risque d'un abaissement du niveau des bacheliers professionnels et de leurs chances en matière d'études supérieures et d'insertion est réel. Au contraire, cette réforme doit pouvoir consacrer le droit à l'erreur de l'élève, tant réclamé par le rapport Calvez-Marcon. Quant à l'idée de développer l'apprentissage en lycée professionnel, c'est une excellente nouvelle, car celui-ci favorisera l'insertion professionnelle des élèves. Je regrette cependant que les conditions de sa réalisation restent floues, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans un contexte de réforme de l'apprentissage qui, bien qu'elle ait apporté des améliorations, comporte encore de nombreuses zones de vigilance, comme le coût de l'apprenti et le reste à charge pour l'employeur, la situation des 32 000 conjoints collaborateurs, qui, n'étant pas salariés, ne peuvent être maîtres d'apprentissage, ou encore, et surtout, le financement des centres de formation des apprentis. Sachant qu'un contrat d'apprentissage sur trois est rompu sur l'initiative de l'apprenti, je regrette que toutes ces réformes ne s'accompagnent pas d'un plan plus global évoquant croissance économique, stratégies de recrutement des entreprises ou encore fonctionnement du monde du travail. Le 17 mai dernier, lors du comité interministériel du tourisme, le Premier ministre a annoncé un grand plan tourisme, défini avec les professionnels du secteur, ayant pour ambition d'ajuster des parcours d'emploi, de faciliter les mobilités et d'adapter les formations aux besoins des employeurs.